La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

L'éligibilité des projets de production ou de stockage de gaz bas-carbone et d'hydrogène bas-carbone aux dispositions dérogatoires ainsi prévues conduirait à une régression du droit de l'environnement pour d'autres filières de production électrique, ce qui ne nous semble pas justifié. Il s'agit donc de restreindre strictement l'application des dérogations aux projets et opérations de production, de stockage

En effet, dans la rédaction actuelle, le périmètre d'application des adaptations prévues aux alinéas 7 à 14 est trop large dans son contenu et imprécis dans sa formulation. Ainsi, alors que le texte prévoit que ces adaptations pourront s'appliquer à la catégorie des « installations industrielles de fabrication ou d'assemblage de produits ou équipements qui participent « qui sont strictement nécessaires ». Les dérogations prévues au I de l'article pourraient également s'appliquer à différents projets de modification industrielle, sans lien avec la transition écologique. Pour éviter les dérives et des situations qui n'auraient pas de pertinence pour lutter contre le changement climatique, le périmètre d'application de cet article doit être strictement restreint aux projets et opérations de production, de stockage ou de transport d'énergie issus

non recyclables, l'utilisation de la chaleur de l'énergie renouvelable et de récupération dans l'industrie et dans les réseaux de chaleur urbains en substitution des énergies fossiles, ainsi que le captage, le stockage et la valorisation de CO2.

aux projets de captage, de stockage et d'utilisation de CO2 dans la liste des installations et opérations concernées par les mesures d'urgence temporaires prévue à l'article

En effet, l'objectif de ces projets est de lutter efficacement contre le dérèglement climatique, comme cela est rappelé dans le compte rendu du conseil des ministres

n° 466 rectifié vise essentiellement à étendre les dispositions aux installations d'utilisation de carbone et de stockage. Or la stratégie nationale ne prévoit pas d'avoir recours massivement à de telles installations,

et, par là même, de garantir davantage de lisibilité aux porteurs de projet, je souhaite soulever la question récurrente du dimensionnement des services administratifs par rapport au flux des demandes. En effet, on constate dans les départements, sur tout le territoire, un manque cruel de moyens humains au sein des services instructeurs. Ce problème a même été de nouveau identifié par le Conseil national de la transition qui, dans son avis sur le projet de loi, indique une « insuffisance des moyens humains et financiers de l'État et des collectivités pour instruire et suivre les projets, et soutenir la structuration de certaines filières d'énergies renouvelables ». Or, sans ces moyens, il est très peu probable probable que nous arrivions à garantir le déploiement accéléré des énergies renouvelables dans le respect de l'environnement et en cohérence avec les spécificités des territoires d'implantation. La réduction des délais d'instruction, dès lors que les services sont sous-dimensionnés dans un secteur en pleine expansion,

tiennent à relever les défis de la transition énergétique sur leur territoire. Ils sont d'ailleurs nombreux à avoir signé des contrats de développement territorial des énergies renouvelables et adopté un schéma départemental des énergies renouvelables.

Cet amendement vise à supprimer l'ajout introduit par la commission d'une période d'un mois durant laquelle doivent être vérifiées la complétude et la régularité d'un dossier de demande d'autorisation pour un projet de production d'énergies renouvelables.

Cet amendement vise à accélérer l'instruction des autorisations environnementales, qui nécessite un meilleur encadrement de la phase de complétude, durant laquelle l'administration demande des compléments aux porteurs de projets.

La phase de complétude est celle au cours de laquelle l'administration demande des compléments aux porteurs de projets, jusqu'à ce que le dossier soit considéré comme complet. Elle constitue donc l'un des moments-clés de la procédure, où nous pouvons gagner en efficacité, sans sacrifier la qualité des dossiers déposés par les porteurs de projets, le respect des normes environnementales ou encore la participation du public.

Pour ce qui est de l'enregistrement, l'étude de complétude dure en moyenne trois mois, alors que le délai est de trois semaines en Suède et de deux mois en Allemagne. Le rapport a donc formulé une recommandation en faveur de l'encadrement de la durée de l'étude de recevabilité, en la portant à un mois à compter de l'accusé de réception du dossier afin de pallier ses défauts et ses carences manifestes. Tel est le sens de cet amendement, qui vise en outre à préciser que l'examen est intégral et que les demandes de complément et correctifs sont regroupées en un seul courrier.

? Cet amendement est pleinement satisfait par le droit en vigueur. Toute demande d'autorisation environnementale est par définition instruite. Le Gouvernement a adressé une circulaire fixant des directives très claires aux préfets s'agissant de l'instruction Nous avons complété ces mesures à l'article 1 par des dispositions dérogatoires pour accélérer notre production d'énergies renouvelables. Par ailleurs, le rejet de la demande d'autorisation environnementale est toujours motivé dans la décision rendue par l'autorité administrative compétente. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle

En effet, il convient d'introduire dans l'étude d'impact des projets éoliens une description de leurs conséquences sur l'eau et les nappes phréatiques, ce qui n'est pas prévu pour ce type d'investissement. La réalisation de ces projets peut nécessiter de creuser le sol en profondeur, ce qui pourrait avoir une incidence sur la qualité de l'eau et les nappes phréatiques.

Je partage votre préoccupation, mon cher collègue, mais l'amendement est satisfait par le droit en vigueur. En effet, le principe de l'étude d'impact, qui découle de l'obligation d'évaluation environnementale des projets, inclut l'eau, l'air, tous les milieux et tous les éléments.

de tenir compte de l'ensemble des impacts des projets. Toutefois, je comprends et je partage vos préoccupations, mon cher collègue. La notion de renouvellement ne fait pas encore l'objet d'une définition législative précise ; un arrêté définit les cas de modification substantielle et notable, ainsi que le régime juridique applicable.

Cet amendement vise à introduire la notion de renouvellement des installations de production d'énergie renouvelable et de ne soumettre à l'examen au cas par cas que les modifications ou les extensions

De plus ce dispositif serait contraire aux dispositions de la directive Projets de 2011, sur l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement, en en excluant certains du champ de l'examen au cas par cas. Le risque de contentieux à l'échelon européen

la mise en place d'une obligation de certification a profité aux quelques gros bureaux d'études nationaux et internationaux, au détriment des experts qui maillent notre territoire. Quel est l'avis de Ces amendements concernent un dispositif inséré en commission, qui vise à améliorer la qualité des dossiers soumis à l'administration pour instruction. Je ne suis pas favorable à la transformation de tout ce qui a été fait en commission en une simple expérimentation. Je suis donc défavorable à l'amendement n°

précise que l'étude d'impact est réalisée sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Il s'agit d'un point fondamental de répartition des responsabilités. L'indépendance entre le bureau d'études et le porteur de projet ne peut donc être le résultat de l'absence de lien contractuel entre eux. Certains maîtres d'ouvrage ont d'ailleurs internalisé une partie des bureaux d'études.

ou scientifiques, les raisons qui l'ont amené à contester l'étude d'impact. Cette clarification permettra au maître d'ouvrage de mieux comprendre la décision de l'autorité.

Avis défavorable.

interne de la directive européenne Projets et la jurisprudence communautaire ont abouti à intégrer, au sein de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, la notion de projet global, l'objectif étant d'éviter un contournement de l'obligation de réaliser une évaluation environnementale en fractionnant artificiellement un projet. Cet article prévoit donc que l'étude d'impact doit porter sur le projet appréhendé dans sa globalité, lorsqu'il est constitué de plusieurs travaux- travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou autres interventions -, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité des maîtres d'ouvrage. Si cette disposition est légitime et pertinente, elle devient complexe en matière d'installations de production d'électricité renouvelable. En effet, les gestionnaires de réseau ne fixent les conditions de raccordement qu'une fois le projet d'installation de production devenu définitif. Cet amendement a donc pour objet de distinguer les travaux de construction, d'installations et d'ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel, qui concernent les installations de production d'électricité renouvelable, des travaux de raccordement, tout en garantissant que chaque projet puisse faire l'objet, le cas échéant, d'une évaluation environnementale et d'une enquête publique.

publique. La même philosophie régit le début de cet article, qui prévoit la désignation de commissaires suppléants, afin de garantir le bon déroulement de l'enquête publique.

le certificat de projet, qui a été généralisé par l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, après avoir fait l'objet d'une expérimentation, dans l'objectif d'accroître la sécurité des porteurs de projets le plus en amont possible des procédures. Ce dispositif permet à tout porteur de projet soumis à autorisation environnementale d'obtenir de la part de l'administration une information complète des régimes de décision et des procédures applicables au projet. Il peut notamment comporter un calendrier d'instruction de la décision, qui peut engager l'administration. Or la commission du développement durable a adopté sa suppression, au motif qu'il aurait été peu utilisé jusqu'en juin 2018, soit un an et demi après son entrée en vigueur. Le certificat de projet ne constitue pas un frein au projet de production d'énergie renouvelable, mais peut faciliter les démarches du demandeur, en lui donnant plus de visibilité. L'allongement des procédures est davantage dû à la partie réglementaire du code, qu'il suffirait de modifier. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l'amendement n° 428. La suppression des certificats de projet

je m'en tiendrai là.

avons réalisé, à la mi-2018, un premier retour d'expérience sur l'utilisation du certificat de projet, une enquête auprès des services déconcentrés. Celle-ci a montré que le certificat avait été utilisé, jusqu'en juin 2018, dans environ 1 % des dossiers soumis à autorisation.

du régime de la participation du public par voie électronique, en lieu et place de l'enquête publique. Nous pourrions le regretter. Il faut rester particulièrement vigilant sur l'importance des enquêtes publiques et de la concertation.

ou d'aménagement, exécutés par des personnes publiques ou privées, qui donnent lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale, après examen au cas par cas.

sur support papier, sur demande ou si le volume et les caractéristiques du projet ne permettent pas la mise à disposition du dossier par voie électronique. Voilà qui paraît suffisant. Ce n'est pas parce qu'il existe une consultation électronique que l'on n'a pas accès aux documents papier. Madame Varaillas,

Considérant que les surfaces d'artificialisation des installations solaires des ouvrages des réseaux publics de transport ou des réseaux de distribution d'électricité sont très faibles et compte tenu des enjeux majeurs de la transition énergétique, il est proposé de considérer ces surfaces comme non artificialisées.

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi Élan, a mis en place la dématérialisation de la réception et de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, codifiée à l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition, qui constitue un progrès pour les demandeurs, s'applique depuis le 1 janvier de cette année aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées dans les communes de plus de 3 500 habitants. Cet amendement vise à étendre cette obligation de dématérialisation à toutes les communes, uniquement pour l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives aux projets de production d'énergie renouvelable. ? La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. En 2018, le Sénat a justement exclu les petites communes du champ de cette obligation,

ne peuvent se faire qu'avec les acteurs locaux, en particulier les élus qui connaissent parfaitement leur territoire. Cet amendement vise à ce que l'autorisation d'exploiter soit non seulement compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie mais aussi avec le document d'orientation et d'objectifs des Scot ou avec certaines orientations d'aménagement et de programmation des PLUi.

L'objet de cet amendement me paraît intéressant, en ce qu'il exige de l'État une plus grande responsabilité dans son rôle de délivrance des autorisations d'exploiter des sites de production d'électricité. Voilà qui correspond à notre intention

À droit constant, la création d'une installation de production d'électricité doit être conforme avec le règlement d'un PLU et doit être compatible avec les orientations d'aménagement de programmation de ce même plan, en application de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme.

PLU, PLUi, cartes communales -aux projets de centrales solaires au sol. Cette disposition n'a pas pour objet de rendre inopposable l'ensemble des règles d'urbanisme. Les projets de centrales au sol devront ainsi toujours respecter les dispositions de la loi Littoral, de la loi Montagne ou des plans de prévention des risques notamment. cet amendement lèverait en réalité toute application des PLU aux projets d'énergie renouvelable pendant deux ans. La commission souhaite que les documents d'urbanisme locaux conservent leur rôle de planification et leur pertinence.

constitue une sérieuse régression environnementale. Cette automaticité ne permet pas l'évaluation de l'opportunité écologique de la réalisation des projets concernés et concurrence différents objectifs environnementaux, notamment ceux de protection de la biodiversité, ainsi que les objectifs de développement que les objectifs de développement durable (ODD), auxquels la France a souscrit. Reconnaître prématurément cette RIIPM à un stade où l'état initial de l'environnement et les impacts du projet ne sont pas encore précisément connus est contraire à l'esprit de la directive Natura 2000, est interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Cet amendement vise donc à supprimer cet article dans son intégralité, afin de maintenir l'évaluation de l'opportunité écologique de la réalisation des projets concernés.

que construire des EnR relève d'un intérêt public majeur, quand il s'agit de préserver la biodiversité, puisque, vous le savez, le changement climatique est l'une des premières raisons d'altération de la biodiversité. En tout état de cause,

d'intérêt public majeur, qui permet de déroger aux interdictions d'atteintes envers certaines espèces végétales ou animales et leurs habitats naturels. Pour en bénéficier, ces installations devaient satisfaire à des conditions techniques définies par décret en Conseil d'État. donc pas d'accorder à n'importe quel projet de production d'EnR la dérogation « espèces protégées » ; l'automaticité de cette raison impérative d'intérêt public majeur était encadrée. En supprimant le décret en Conseil d'État, la commission a fortement assoupli les conditions de cette RIIPM appliquée aux projets d'installations de production d'énergies renouvelables. ne seraient plus seulement concernés les grands projets permettant de garantir la sécurité d'approvisionnement énergétique qui, pour cette raison même, pouvaient bénéficier du caractère de RIIPM,

d'autre part, nous estimons nécessaire que les conditions que doivent satisfaire les projets d'EnR soient également fixées en s'assurant de la capacité de notre outil de production à préserver notre souveraineté industrielle. L'amendement Cet amendement vise à indiquer que la reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public majeur est précisée par décret en Conseil d'État. À première vue, il peut sembler similaire aux deux amendements

d'électricité et d'électrons dans les tuyaux

Il convient donc de bien tenir l'objectif de décarbonation. Il serait dommageable que le développement précipité, dans l'ensemble du territoire, de projets EnR intermittents mal évalués, accroisse notre dépendance aux énergies fossiles et compromette notre stratégie de décarbonation.

D'abord, cette mesure n'a rien à voir avec l'objet du projet de loi, à savoir l'accélération de la production des énergies renouvelables. Prévoir que la DUP puisse valoir reconnaissance du caractère d'opérations

Pis encore, ces dispositions sont contraires à l'objectif de valeur constitutionnelle « d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi », pour citer le Conseil constitutionnel. Ensuite, cette mesure est contraire au droit européen.

lorsqu'elles apprécient le bien-fondé d'une dérogation, les autorités nationales doivent se demander si elle est justifiée par l'une des raisons figurant à l'article 16 de la directive. Il y a lieu également de considérer le type et l'importance de la raison, par rapport à l'intérêt de l'espèce protégée dans les circonstances spécifiques concernées afin de déterminer si la dérogation est opportune. Le projet de loi prévoit d'entériner l'opportunité d'un projet d'EnR en amont de la connaissance effective des espèces auxquelles il portera atteinte. L'objet de cet amendement est donc de limiter la possibilité accordée par cet article aux seuls

Mme la ministre. examinée par le juge dans le cadre d'un contentieux. Il s'agit bien d'une notion distincte, nettement plus restrictive, de celle de déclaration d'utilité publique. Le dispositif proposé dans cet article doit permettre de stabiliser le critère de raison impérative d'intérêt public majeur, dès la déclaration d'utilité publique, pour les opérations reconnues d'utilité publique nécessitant, en outre, une dérogation « espèces protégées ». Contrairement à ce qui est indiqué dans l'objet de cet amendement, le III de l'article 4 ne prévoit pas la reconnaissance automatique de la raison impérative

un projet peut être reconnu comme répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur ou si, au contraire, il ne présente pas les garanties suffisantes pour l'être. Le renvoi à un décret en Conseil d'État prévu par le projet de loi permettra au pouvoir réglementaire de fixer les conditions de procédures

La reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public majeur permet de contourner un certain nombre de règles ; il est donc essentiel d'en encadrer l'attribution. Au-delà des conditions techniques, la raison impérative d'intérêt public majeur devrait être appréciée au regard de la quantité d'énergie produite et de l'ampleur de l'atteinte à la biodiversité, tout en tenant également compte de la participation du projet concerné à la réalisation des objectifs régionaux de production d'énergies renouvelables.

Les énergies renouvelables doivent être développées, mais pas n'importe comment ni à n'importe quel prix. Une approche plus nuancée et équilibrée doit être retenue. Quel est l'avis de

de rendre plus explicite la conservation de la déclaration d'utilité publique d'une canalisation existante convertie pour transporter de nouveaux produits, tels que l'hydrogène, visant à l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone, tout en garantissant la participation du public, dans le respect des principes généraux du code de l'environnement.

De plus, la demande d'autorisation d'exploiter étant soumise à des autorités qui peuvent être différentes de celles ayant lancé la procédure de mise en concurrence,

omis quelques éléments techniques ou administratifs à régulariser plus tard, et sans interrompre nécessairement l'intégralité d'un chantier litigieux. Le juge doit motiver le refus de surseoir à statuer, ce qui ajoute une une contrainte influant sur sa décision. Les ajouts prévus par la commission font également peser une pression supplémentaire sur les requérants, qui ne sont pas toujours en capacité d'affronter les procédures judiciaires, toujours impressionnantes pour la majorité de nos concitoyens.

voire bancals. Il nous semble donc nécessaire de supprimer l'article 5 pour permettre une instruction des dossiers, y compris judiciaires, sans dérogation particulière.

autorisation environnementale. Or le juge dispose déjà de ce pouvoir de régularisation. Cette disposition comporte un risque : si l'on poursuit l'exécution d'une décision environnementale sans attendre que la procédure qui aurait dû mener à cette autorisation soit correctement mise en oeuvre, des dégâts irrémédiables peuvent être causés. La régularisation pourrait conduire à ce que des mesures d'évitement ou de réduction des impacts soient prescrites dans le cadre du bon déroulé de la procédure. Si les travaux ont déjà eu lieu, il sera trop tard pour mettre en oeuvre ces prescriptions. C'est pourquoi cet amendement vise à compléter cette disposition en prévoyant que le sursis à statuer soit obligatoirement accompagné d'une suspension de l'autorisation, pour éviter que des travaux soient poursuivis en méconnaissance de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) qui pourrait être identifiée lors de la régularisation.

les dispositions de l'article 5 s'appliqueront aux contentieux en cours, et non pas à ceux qui naîtront après la publication de la loi. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat ... une sagesse plutôt favorable

Monique de Marco. L'autorisation environnementale permet de simplifier et d'accélérer un certain nombre de procédures administratives et juridiques. Elle permet également de sécuriser des porteurs de projet. lorsqu'une partie de cette autorisation est annulée ou fait l'objet d'un sursis à statuer, le porteur de projet est confronté à de nombreuses incertitudes. En effet, continuer les travaux engagés sans attendre la fin de la procédure de régularisation peut se révéler dommageable. Le chantier de la déviation de Beynac, en Dordogne, et sa suspension par le Conseil d'État doivent nous servir d'exemple. Trop d'argent public a été gâché pour un projet qui a finalement été suspendu dans son intégralité

font l'objet d'un recours. Bien que le droit à un recours effectif soit légitime, il est utilisé à outrance par certains et semble parfois relever davantage d'une tentative d'obstruction pour empêcher certains projets de voir le jour. Même si des mesures législatives et réglementaires ont été introduites par le projet de loi aux fins de réduire les délais de traitement des contentieux, il est dorénavant nécessaire de réduire à la source les recours abusifs. C'est pourquoi cet amendement vise à introduire un dispositif de sanction des recours abusifs contre les autorisations environnementales, titre I du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement.

vise donc à rendre le dispositif opérationnel d'un point de vue juridique, en précisant que l'adhésion au fonds doit être réalisée entre la délivrance de l'autorisation et le lancement des travaux. Cela permet de ne pas créer de régime dérogatoire au droit commun dans les projets de construction. Cet amendement a également pour objet de rendre l'adhésion au dispositif optionnelle pour les producteurs lauréats d'un appel d'offres ou d'un complément de rémunération obtenu par arrêté tarifaire.

pourquoi il nous a semblé essentiel d'assurer une meilleure couverture de ce risque en créant, à l'article 5 , un fonds de garantie. Nous nous réjouissons que le Gouvernement se saisisse de cette proposition importante, en coconstruisant à partir du dispositif prévu par la commission. Je précise que ce fonds de garantie a été plutôt bien accueilli par l'ensemble des acteurs et des opérateurs du secteur.

se rapportant aux cotisations fournies par les entités publiques qui financent le fonctionnement des opérateurs producteurs d'énergie. il ne faudrait pas que ces entités publiques viennent compenser les pertes éventuelles enregistrées par les opérateurs. Il s'agit donc d'une précaution que nous préférons intégrer d'emblée dans le texte. Quel est l'avis

au Président de la République de décider seul par voie d'ordonnances. Si certains raccordements de travaux doivent être faits dans les plus brefs délais, il convient que les autorités compétentes bénéficient des moyens adéquats pour se saisir de l'urgence et entament les procédures nécessaires au bon fonctionnement des réseaux.

n'est pas souhaitable, pour plusieurs raisons. D'une part, tous les acteurs qui ont été interrogés- élus locaux, professionnels, gestionnaires -sont largement favorables à cette habilitation, qui, je le rappelle, porte sur une matière très technique pour des procédures dérogatoires est constitutionnellement justifié. Sans une simplification de nos procédures de raccordement, il est illusoire d'espérer atteindre nos objectifs de transition énergétique !

Il est donc essentiel de consulter ceux qui vivent sur les territoires concernés afin de garantir l'acceptabilité sociale de ces ouvrages. Nous ne pourrons atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables si nous n'arrivons pas à convaincre la population. Un affaiblissement quantitatif et qualitatif de la consultation du public ne ferait qu'alimenter les recours et les oppositions aux projets, d'autant que rien ne justifie un allégement des modalités de consultation. Un rapport de 2021 du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) souligne que la durée des procédures n'est pas la cause déterminante des délais de mise en oeuvre. Aussi, réduire la consultation du public en légiférant par ordonnances serait contre-productif. Quel est l'avis de

la modification des conditions de participation du public est une demande forte des acteurs économiques, afin de simplifier et d'accélérer les raccordements aux réseaux de distribution et de transport d'électricité.

économiques, a pour objet d'ajouter la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à la liste des acteurs associés à l'élaboration de l'ordonnance sur la simplification et l'accélération des procédures de raccordement aux réseaux publics de distribution et de transport d'électricité.

de rapport n'est pas opportune. Tout d'abord, le Sénat est par principe opposé à de telles demandes. Ensuite, il serait curieux de demander un rapport sur le raccordement, alors qu'une réforme d'ampleur est prévue sur le sujet par l'habilitation à légiférer par ordonnances mentionnée à l'article 6. Enfin, sur le fond,

Cette opacité nous inquiète. On sait en effet que des investissements importants seront nécessaires pour permettre une plus grande flexibilité et une sécurité d'approvisionnement sur les réseaux, ainsi que le raccordement de capacités de production intermittentes. Lorsqu'un opérateur d'énergies pilotables construit un aménagement, il doit prendre en charge les frais de raccordement. Pour les EnR toutefois, il n'y a pas de parallélisme, alors même que ces opérateurs sont prioritaires sur le réseau et que les coûts de raccordement, par exemple pour les parcs éoliens en mer qui nécessitent des raccordements lourds, sont particulièrement importants. On nous dit que les dispositions des articles 6 et 6 doivent clarifier l'identification des utilisateurs, la prise en charge par le Turpe d'une partie des coûts de raccordement et la création d'un forfait raccordement, dont, franchement, on n'apprend pas grand-chose à la lecture du projet de loi, et ce tout en inscrivant dans la loi la suppression de la contribution de certaines collectivités au financement de l'extension du réseau À la lecture de ces articles, il est impossible de savoir quelle sera la part payée à l'avenir par les producteurs et si elle permettra bien de couvrir une part des investissements faits par les gestionnaires de réseaux. De même,

? La commission a souhaité inscrire directement dans la loi certaines dispositions de l'habilitation à légiférer par ordonnances : la suppression de la contribution des communes ou de leurs groupements au financement de l'extension des réseaux de distribution d'électricité, ainsi que l'octroi à la CRE d'une compétence pour approuver les contrats d'accès aux réseaux de distribution et de transport d'électricité. Ces inscriptions dans le « dur » de la loi concourent à borner le champ d'action du Gouvernement. Si, tout

La première partie de l'amendement vise à modifier, sur la forme uniquement, la rédaction de l'article 6 relative à l'approbation des contrats d'accès au réseau par la Commission de régulation de l'énergie. La seconde partie apporte des évolutions attendues au dispositif des S3REnR, tout en ne revenant pas sur les grands principes de ces derniers, à savoir la planification du déploiement du réseau et la mutualisation des ouvrages auxquels sont attachés les acteurs consultés. Ces évolutions sont destinées à rationaliser les phases d'élaboration des schémas de planification des réseaux, notamment en fiabilisant les gisements pris en compte pour l'élaboration des schémas. Les modifications proposées tendent également à renforcer la portée anticipatrice des schémas en fixant un horizon de dix à quinze ans pour ceux-ci et en prévoyant que certains ouvrages jugés sans regret pour la collectivité puissent être lancés dès la validation du schéma. Enfin, l'amendement a pour objet que les travaux de raccordement au réseau électrique et de pose de fibre optique puissent être mutualisés pour accélérer la mise en service des installations et optimiser les coûts

de la contribution communale au réseau d'électricité et l'harmonisation des contrats d'accès au réseau de distribution d'électricité sont maintenues et même complétées, puisque cette harmonisation est étendue par l'amendement au réseau de transport d'électricité. Plus encore, les dispositions relatives au modèle de contrat ou aux méthodes de coûts, de même qu'au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, consistent essentiellement en des recodifications. Enfin, certaines novations sont positives pour nos professionnels l'allongement de cinq ans de la durée du S3REnR, l'institution d'un tel schéma en Corse, l'exonération des installations de petite puissance de contribution et l'accès non discriminatoire aux réseaux. Je relève que ces dispositions offrent aussi une possibilité de coupler les travaux de raccordement en matière d'énergie avec ceux qui sont réalisés en matière de fibre optique. Sur ce point, elles consistent en la reprise d'une disposition que le Sénat avait fait adopter, sans réussir à la faire prospérer, dans le cadre de la loi Asap de 2020, sous l'égide de notre rapporteur d'alors, Daniel Gremillet. C'est un hommage tardif, mais bien réel à son travail, qui a été fort apprécié ! J'ajoute que j'ai veillé à ce qu'aucune disposition bouleversant les conditions financières

de notre groupe. Les réseaux intérieurs des bâtiments (RIB) ont été introduits par l'article 16 de la loi du 30 décembre 2017. Ce mécanisme doit inciter les promoteurs immobiliers et les foncières à investir dans la construction de bâtiments vertueux, en produisant leur propre électricité sur site, ce qui favorise le développement des énergies renouvelables. La rédaction actuelle est néanmoins limitée aux seuls immeubles de bureaux, excluant tout bâtiment tertiaire mixte, ce qui conduit dans la pratique à un accroissement relativement faible de ce type d'investissement. Il apparaît donc essentiel d'élargir le bénéfice de cette mesure, en intégrant toute la diversité des usages des entreprises occupantes au sein d'un même bâtiment, sans la limiter aux seuls espaces de bureaux, afin que les propriétaires de bâtiments tertiaires comprenant des parcs de stationnement extérieur concernés par l'article 11 soient directement et rapidement incités à la réalisation de ces ouvrages. Cet élargissement maîtrisé de la notion de réseau intérieur permettra, au lieu de revendre au réseau l'électricité produite sur site, de favoriser l'autoconsommation de celle-ci dans le cercle limité des entreprises occupant l'ouvrage, qui pourront ainsi accéder à une énergie verte à un coût limité pour au moins une partie de leur consommation.

qui sont des réseaux privés d'électricité permettant des mutualisations entre bâtiments professionnels. La commission a déjà autorisé par le passé des élargissements, y compris récemment dans la loi Climat et résilience de 2021. L'ajustement prévu au travers de l'amendement est raisonnable, car il ne s'agit que de prévoir que les bâtiments faisant l'objet d'un RIB puissent être

En effet, une loi de 2017 a permis de sécuriser juridiquement les RIB comme schémas de distribution d'électricité dans les immeubles de bureaux appartenant à un propriétaire unique. L'objectif était de s'adapter à la spécificité de l'occupation de ces immeubles, qui connaissent, par exemple, des changements de locataires fréquents, tout en encadrant la possibilité de recourir à ce type de schéma pour ne pas remettre en question le principe général selon lequel ce sont les gestionnaires de réseau public qui acheminent l'électricité produite jusqu'au consommateur final. En ouvrant la possibilité de raccorder à un réseau intérieur, c'est-à-dire à un réseau privé, tout type d'installation de consommation dès qu'il y a une entreprise tertiaire dans l'immeuble,

L'article 7 prévoit de faciliter l'installation de panneaux photovoltaïques sur les délaissés routiers et autoroutiers. L'idée de valoriser des terrains inexploitables au milieu de bretelles ou d'embranchements de voies est bien sûr excellente. Une question reste cependant en suspens, après l'étude d'impact et l'avis du Conseil d'État, qui ne se concentrent que sur la production d'énergie de ces panneaux. Quel est l'impact sur les contrats de concession de la valorisation de ces terrains et des futures installations ? En effet, alors que les contrats de concession sont censés pour la grande majorité prendre fin entre 2032 et 2036, les autoroutiers font tout pour voir les contrats prolongés, notamment en invoquant des investissements non prévus à l'origine, tels que ceux qui permettent le déploiement de bornes électriques ou des énergies renouvelables. Dès lors, ne risque-t-on pas d'ouvrir la boîte de Pandore ? Madame la ministre, pouvez-vous nous rassurer sur cet impact avant que nous n'entamions l'examen de l'article ? Le verdissement des autoroutes est une nécessité. faut aussi mettre fin à des contrats de concession qui sont particulièrement déséquilibrés, comme l'a démontré la commission d'enquête sénatoriale de 2020.

étend la dérogation au principe d'inconstructibilité prévue par l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme à l'ensemble des espaces situés le long des autoroutes et des grands axes routiers, pour permettre l'installation de projets de production d'énergie solaire. Néanmoins, il se trouve que cette dérogation n'est pas possible sur l'ensemble de notre territoire. En effet, certains PLU comprennent des interdictions aux abords des routes ou autoroutes qui sont opposables aux projets solaires. Cela constitue donc un frein, alors que ces terrains, souvent inutilisés, pourraient être mobilisés. C'est pourquoi cet amendement vise à préciser que cette dérogation est applicable automatiquement, nonobstant toute disposition contraire des PLU.

pourrait favoriser le changement d'affectation de terres agricoles. En effet, de nombreuses terres agricoles se trouvent à proximité de routes ou d'autoroutes, notamment dans les départements très urbanisés. Le présent amendement vise donc à empêcher le changement d'affectation de terres agricoles pour permettre l'installation de projets de production d'énergie solaire. Cabanel. Il s'agit d'un amendement de repli, qui tend à empêcher le changement d'affectation de terres agricoles pour permettre l'installation de projets d'énergie renouvelable.

l'étude d'impact ne comporte aucun chiffrage. Nul doute que le potentiel est important. Nous sommes inquiets du risque que cela représente pour les terres agricoles qui longent les routes de notre pays,

pour les routes à grande circulation. Il tend à préciser que les infrastructures concernées par la levée de l'interdiction de construire sont celles qui n'affectent pas

de publicité. Or ce projet de loi permet l'implantation d'installations solaires le long des grands axes routiers, quels que soient leur nature, leur qualité et leur propriétaire. L'interdiction de construction aux abords des routes à grande circulation, qui date de 1995, avait bien pour objet d'inciter les collectivités à engager une réflexion préalable pour améliorer l'aménagement des abords des routes, notamment en entrée de ville. Notre amendement tend donc à préserver, et même à conforter, les efforts réalisés par les communes en vue d'améliorer et de préserver la qualité urbaine, architecturale et paysagère de nos entrées de villes.

sont contraires à l'esprit de l'article 7, qui lève une contrainte législative à l'installation des panneaux solaires en bord d'autoroutes ou de routes nationales, mais qui laisse la possibilité aux élus locaux, dans le cadre de leurs documents d'urbanisme, d'encadrer ces installations.

production d'énergie solaire qui n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol et qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées.

puisque l'article 7 ne dessaisit pas de leurs compétences les autorités compétentes en matière d'urbanisme. Autrement dit, si un document d'urbanisme prévoit des restrictions d'installation, ces restrictions seront toujours valables, malgré l'assouplissement permis par l'article. L'avis de la commission

est à M. Patrick Chauvet. Dans la mesure où l'installation des infrastructures de production d'énergie solaire sur les terrains des communes et des EPCI situés le long des grands axes routiers sera facilitée, il est indispensable de permettre aux élus locaux de s'assurer de la cohérence des installations envisagées avec, notamment, la trajectoire du ZAN qu'ils doivent désormais respecter. C'est d'autant plus important lorsque c'est l'EPCI qui est compétent en matière d'autorisation d'urbanisme et lorsque les communes sont couvertes par une carte communale ou le règlement national d'urbanisme (RNU).

Mme Marie-Claude Varaillas. Par cet amendement, nous souhaitons profiter de l'exemple montré par l'État, avec l'article 8, pour proposer également le déploiement d'installations de produits d'énergies renouvelables sur les espaces appartenant à des à des entreprises publiques ou privées. Nous avons ciblé les entreprises de plus de 250 salariés, car nous avons estimé que cette catégorie pouvait disposer d'espaces bâtis plus importants que les catégories inférieures. Il s'agira de remettre une étude financée par les entreprises elles-mêmes, mais qui pourra contribuer à les aider dans le développement de sites de production sur les espaces leur appartenant. Ce sont aussi ces entreprises qui savent le mieux quels espaces peuvent, ou non, être valorisés, même si le préfet, le référent unique prévu par cette loi, aura à coeur de proposer des installations sur les espaces repérés. Je pense par exemple à la SNCF, à La Poste ou à d'autres grandes entreprises nationales qui disposeraient d'un patrimoine foncier propice à ce type d'installations. Nous en connaissons tous dans nos départements. Nous profiterons ainsi des espaces déjà artificialisés pour soutenir le déploiement du site de production, y compris sur des espaces non accessibles au public. Quel est l'avis de la

ou d'hydrogène renouvelable sur les friches, au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme, ou sur des stocks de saumures. Bien que certaines dérogations puissent paraître légitimes sur les sites très dégradés, où il est impossible d'entreprendre une activité en en raison de la toxicité des lieux, celle qui est instaurée par l'article 9 est trop large. En effet, en l'absence d'activités humaines, que ce soit dans des friches industrielles ou sur d'anciens terrains militaires, la nature reprend ses droits. Des espèces réinvestissent ces lieux, qui présentent des habitats favorables, des sites de repos et d'alimentation, des reposoirs, voire des habitats protégés au titre de la directive Habitats. Par conséquent, cette définition très large- la plupart des sites nécessitent un réaménagement ou des travaux avant réemploi -risque de conduire à investir des lieux qui abritent des sites présentant des enjeux de biodiversité. Le projet de loi prévoit une étude pour démontrer que le projet n'est pas de nature à porter atteinte à la biodiversité,

l'objet de l'amendement n° 73 rectifié, la dérogation à la loi Littoral permise par l'article 9 du projet de loi n'est pas trop large : elle est au contraire très encadrée, avec un avis obligatoire de la commission départementale de la nature, la nature, des paysages et des sites. Je rappelle également que l'autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l'environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d'incident ou d'accident. Je rappelle enfin qu'il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d'installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d'intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. La dérogation, j'y insiste,

L'objet de cet amendement est de rétablir l'article 9 dans sa rédaction initiale, en l'adaptant pour tenir compte des débats en commission. L'amendement vise à permettre un équilibre entre les enjeux liés à la préservation des espaces littoraux et le développement des énergies renouvelables. En effet, le texte adopté en commission conduit à admettre une dérogation à la loi Littoral dont le champ est considérable, ce qui nous semble fragiliser la constitutionnalité de la mesure. Il convient de le rappeler, le Conseil constitutionnel exerce, depuis deux décisions de 2017 et 2018, un contrôle sur les adaptations de la loi Littoral au regard de la Charte de l'environnement. Il veille donc à ce que les dérogations soient strictement proportionnées. C'est la raison pour laquelle le dispositif doit demeurer équilibré et limité, au risque d'être entièrement censuré par le Conseil constitutionnel en cas de saisine, ce qui n'est pas notre objectif. Dans ce contexte, l'emploi du terme « friches » présente tout son intérêt, en ce qu'il permet de s'appuyer sur une notion désormais définie définie dans le code de l'urbanisme, à la suite de l'adoption de la loi Climat et résilience. Cela permet d'éviter les difficultés d'interprétation que poserait le recours à la notion de sites dégradés, qui n'est pas définie par les textes. Cette notion permet déjà d'englober une grande variété de sites, tels que les espaces déjà artificialisés, les anciennes carrières ou encore les anciennes décharges. Elle est donc susceptible d'inclure un grand nombre de sites dégradés, sans qu'il soit besoin de viser expressément cette notion aux contours imprécis. le texte adopté en commission conduit également à étendre le dispositif à d'autres types d'ouvrages, dont les installations solaires thermiques, les installations de stockage d'énergie et les installations d'hydrogène bas-carbone.

à minimiser l'impact paysager. Enfin, il convient de préciser que les collectivités seront associées au processus d'élaboration du décret fixant les sites concernés par le dispositif. mention de la consultation obligatoire du maire ou, le cas échéant, du président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme n'est en revanche pas utile, puisque cette

Nous avons déjà eu ce débat lors de l'examen de la loi Climat et résilience, puis, de nouveau, lors de l'examen de la proposition de loi visant à permettre l'implantation de panneaux photovoltaïques sur des friches, déposée par notre collègue Didier Mandelli et adoptée à l'unanimité par le Sénat le 22 février 2022. Sur le principe, nous partageons l'objectif de reconversion des friches, mais nous demeurons vigilants quant à la préservation des espaces littoraux. C'est la raison pour laquelle notre amendement vise à limiter les installations de production d'énergie solaire à la vingtaine de friches identifiées, que nous avons déjà évoquées.

Notre objectif est d'assurer la cohérence entre, d'une part, les actions de prévention, de sauvegarde et de restauration programmées sur l'espace littoral, et, d'autre part, les éventuels projets d'implantation d'équipements photovoltaïques, ce que nous avions également unanimement approuvé lors de nos travaux, voilà un peu plus de six mois.

ce dernier] à donner un avis sur le décret qui listera[it] les friches dans lesquelles la dérogation à la loi Littoral aura[it] vocation à s'appliquer. C'est la raison pour laquelle cette concertation a[vait] été retirée. Si elle [avait été] maintenue, elle [aurait nécessité] de modifier

anciens périmètres de protection de captage d'eau et ouvrages de captation d'eau de pluie. Or ces dernières zones étant souvent naturelles, il ne nous paraît pas

entend par " friche " tout bien [ ...] inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables